et Alexandre Basquin, qui a remplacé notre ancien collègue Éric Bocquet. Au nom du Sénat, je leur souhaite la bienvenue. L’ordre

pleuré Thomas, le Rugby Club Romanais Péageois pleure Nicolas. Thomas Perotto a été poignardé lors du bal de Crépol ; Nicolas Dumas a été victime d’une fusillade à l’entrée de la discothèque Le Seven, à Saint Péray. Combien de jeunes sont victimes de mort violente depuis un an ? Si l’on ne regarde que la semaine dernière, les faits ayant conduit à la mort violente de jeunes gens sont en croissance exponentielle.

Les morts s’enchaînent à une cadence infernale. Le mois dernier, c’était à Marseille et à Nevers que les morts se succédaient. Nous avons bien évidemment une pensée pour toutes ces victimes et pour leurs familles, leurs amis. Mais la compassion ne suffit pas, ne suffit plus. En ce moment, une marche blanche démarre à Romans sur Isère. Cette ultraviolence se développe dans les villes médianes, à la campagne, même si les villes ne sont pas épargnées, comme le démontre l’attaque à la hache dans le RER lundi matin. Face à des comportements de plus en plus violents et de plus en plus extrêmes, dans une société où la violence devient quotidienne et quasiment banale, que compte faire le Gouvernement pour que nos enfants et nos petits enfants puissent se promener, participer à la vie associative, s’amuser, étudier, travailler, bref, vivre en toute sécurité ce que je trouve le plus difficile, c’est d’être soumis à cette chronique, malheureusement devenue trop banale, d’événements abominables. Et je suis surpris par ce rajeunissement, cet effroyable rajeunissement

quelles que soient nos étiquettes et nos appartenances politiques. Je pense que, sur une cause aussi importante, nous devons nous rassembler. Et, je n’en doute pas, nous nous rassemblerons. Monsieur le ministre, il y a effectivement une insécurité réelle au quotidien. La sécurité au quotidien ne peut pas se décréter ; il faut la vivre. Nous en avons tous besoin, et nous l’attendons avec impatience. Luttons sans faiblesse contre l’insécurité, mais sans démagogie, et dans le respect de l’État de droit. Vous nous trouverez pour avancer ensemble, afin de mettre fin à ce fléau qui gangrène notre vie. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. Mille deux cent

À Cholet, l’usine était implantée depuis 1970. C’est dire le nombre de générations qui y ont travaillé, l’attachement de la population et le traumatisme pour tous ces salariés et pour les familles. Mon premier message aujourd’hui sera donc pour exprimer notre soutien

Nous avons exprimé notre exigence, dans un contexte difficile pour la filière automobile, en particulier pour les activités de pneumatiques de Michelin, d’un accompagnement des salariés qui soit exemplaire. exemplaire, cela signifie apporter une réponse personnalisée, afin qu’aucun salarié ne reste sur le bord du chemin. Cette première exigence se double d’une exigence à destination des territoires. Redynamiser et réindustrialiser le territoire, c’est l’engagement qu’a pris la direction de Michelin.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, au nom de notre groupe, je tiens à exprimer notre immense solidarité à l’égard de nos voisins espagnols. Gardons en mémoire toutes celles et tous ceux qui ont péri noyés. écologique, Jean François Rapin et moi même vous avons remis voilà quelques semaines notre rapport parlementaire consacré à la prévention des inondations en France. Nous savions que le péril était grand et sans doute sous estimé.

Évoluer, faire preuve de solidarité, mener des politiques de prévention et de résilience massive, simplifier : ce sont les actions que nous attendons. Madame la ministre, je souhaite insister ici sur un objectif, celui de la bonne gestion de nos cours d’eau. Car oui, mes chers collègues, nous allons devoir considérablement simplifier le bon entretien des cours d’eau affectés par des débordements ! Oui, nous allons devoir mieux anticiper les inondations en renforçant nos procédures d’alerte. Oui, nous allons devoir réformer très vite la Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention Oui, nous allons devoir engager des concertations avec nos agriculteurs pour parvenir à des pratiques agricoles plus adaptées pour l’écoulement des eaux ! Oui, nous allons devoir aménager et reconstruire autrement, sans trembler

Vous évoquez la gestion des cours d’eau. Vous le savez, dans le Pas de Calais, nous avons expérimenté un certain nombre de simplifications. Elles ont porté leurs fruits, permettant de gagner jusqu’à sept mois dans l’exécution des travaux. Vous même, qui avez

et Républicain. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur. Plus personne n’ignore désormais que le narcotrafic menace les intérêts fondamentaux de la Nation. La commission d’enquête du Sénat en a démontré au printemps la violence criminelle, l’emprise territoriale, la puissance financière corrosive. sceaux allez faire des annonces à Marseille. J’ai compris que nous aurions le débat dans cet hémicycle au mois de janvier. Notre groupe prendra toute sa part à cet effort répressif, indispensable et urgent. Ma question concerne le dernier kilomètre du trafic, c’est à dire ce qui se passe dans nos métropoles, dans nos villes, dans nos villages. Les maires n’ont jamais autant fait pour la sécurité, avec 33 % d’augmentation des polices municipales. Pourtant, ils sont parfois mis au banc des accusés. En réalité, ils Faire peser sur les maires une responsabilité centrale dans de tels drames constitue un bien mauvais procès. Le Congrès des maires consacrera d’ailleurs pour la première fois une table ronde au narcotrafic. Vous l’avez vu, à Rennes, à Poitiers, à Nîmes, nos élus, qui sont en première ligne, attendent un soutien puissant de l’État. Dans un esprit d’union nationale, nous le leur devons. Monsieur le ministre, quelles sont vos pistes de travail ?

Monsieur le ministre, je note avec satisfaction de nombreux points de convergence. Ceux ci n’effacent pas des divergences sur d’autres points,

alors même que le groupe, appartenant à la huitième fortune de France, a réalisé 33 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, qu’il a versé près de 300 millions de dividendes entre 2022 et 2023

Et, malgré cela, encore une fois, ce sont les salariés qui vont payer la note des erreurs stratégiques des dirigeants d’Auchan, le tout sans réelle réaction des pouvoirs publics.

Cette réponse ne nous convainc pas. Elle n’est pas à la hauteur des enjeux. Les 3 000 salariés qui risquent de perdre leur emploi, de même que l’ensemble des contribuables,

d’autant que le risque d’un plan de restructuration beaucoup plus important n’est pas à exclure ? Au delà, va t il enfin accepter une véritable conditionnalité des aides publiques au renforcement de l’information des salariés quant à l’usage qui en est fait et au contrôle du juge ? La

Ces employés, dont le savoir faire et l’engagement contribuent à la renommée de l’entreprise, se retrouvent aujourd’hui dans une incertitude professionnelle totale. Derrière les chiffres, il y a des familles, des parcours de vie et un patrimoine industriel local qui risque de disparaître ; mon collègue Emmanuel Capus l’a très bien expliqué tout à l’heure. Que pouvons nous faire pour que le même scénario ne se reproduise pas demain, que ce soit à Troyes, à Blavozy, en Haute Loire, ou ailleurs en France ? Aujourd’hui, c’est toute la filière automobile européenne qui est menacée de déclassement. En France, c’est Michelin, le leader mondial du pneu, qui chancelle. En Allemagne, c’est Volkswagen, constructeur emblématique et figure de proue de l’industrie, qui flanche. En Suède, c’est le fabricant de batteries Northvolt qui est au bord de la faillite. En réalité, c’est l’ensemble de la filière automobile mondiale qui doit faire face aujourd’hui à une véritable révolution industrielle et à un changement radical de paradigme. Dans ce contexte global, la compétitivité de la filière européenne est sérieusement en difficulté à cause d’une réglementation excessive, d’un coût de l’énergie élevé et d’une concurrence déloyale du mastodonte chinois. Nous sommes à un tournant majeur de l’avenir de notre filière automobile. Il nous faut dès à présent préparer cette mutation si nous voulons empêcher la crise de remonter toute la chaîne de valeur. Cette phase de transition ne doit pas être une phase de déclin fatal. Michelin s’est engagé à créer au moins autant d’emplois que ceux qui seront supprimés. Je le salue. Mais, plus globalement, il est urgent d’accompagner ces mutations inévitables. Il faut conclure ! La mise en place d’un plan national de restructuration est nécessaire pour s’assurer que la transformation se fasse chez nous,

nous avons besoin d’une Europe forte. Plus que jamais, nous avons besoin d’une France forte dans l’Europe.

Il y a un peu plus d’un an, le président Aliyev menait une opération militaire d’épuration ethnique des populations arméniennes du Haut Karabagh. Le Sénat avait dénoncé le régime d’Aliyev, il avait demandé des sanctions. Loin de calmer le président Aliyev, l’organisation de la COP29 le pousse à exacerber la répression contre les populations arméniennes, à menacer toujours plus l’Arménie et à enfermer les opposants politiques. Madame la ministre,

Fusillades à Valence et à Rennes, bus incendiés, barbecue sauvage dans la métropole de Lyon, attaque à la hache dans le RER : de nombreux faits divers ont défrayé la chronique ces derniers temps.

Plus généralement, nous sommes nombreux à nous interroger sur les causes profondes de cette dégradation et sur les moyens de l’enrayer. Citoyens, élus locaux, nous ne pouvons plus assister impuissants à ce déferlement de haine et de violence. Le constater et le déplorer est une chose ; agir et le combattre en est une autre. Quels moyens déploierez vous pour rétablir la sécurité publique ? De quel arsenal pénal disposez vous ? Comment aider les élus locaux à rassurer leurs administrés ? Il faut stopper l’hémorragie et s’attaquer aux causes profondes. La seule chose qui permet au mal de triompher est l’inaction. Monsieur le ministre, nous connaissons votre courage, et nous comptons sur votre détermination.

les causes du mal. Elles sont profondes, et le mal vient de loin. J’en citerai deux. La première, c’est que lorsque, en 1968, on a dit qu’il fallait « interdire d’interdire », on a fait beaucoup de mal à la société. Cette permissivité a fait beaucoup de mal.

moi, détruit les liens entre tous et affaiblit tous nos cadres communs, au point que de jeunes individus n’éprouvent même plus de sympathie les uns pour les autres, les bandes et les groupes étant structurés uniquement par une sorte de charisme de la violence.

L’effroyable attaque terroriste du 7 octobre 2023 par le Hamas – rappelons le, quarante huit de nos compatriotes y ont péri – et la riposte d’Israël qui s’est ensuivie ont de lourdes conséquences en France, notamment dans les établissements d’enseignement supérieur.

Les partenariats internationaux des établissements d’enseignement supérieur constituent pour la France un bel outil de rayonnement intellectuel, scientifique et culturel dans le monde. le comportement de certains étudiants, leurs dérives et leurs initiatives poussant à la suspension de partenariats internationaux pourraient dégrader l’image de notre enseignement supérieur et affaiblir le rayonnement international de la France. Monsieur le ministre, quelles réponses apporterez vous face à cette situation ?

vous m’interrogez sur la motion adoptée par le conseil d’administration de Sciences Po Strasbourg, sur une décision du président de Sciences Po Paris, et plus généralement sur les conséquences de telles initiatives sur le rayonnement de nos établissements à l’étranger. En ce qui concerne Sciences Po Strasbourg, j’ai souhaité réagir sans délai

concerne Sciences Po Paris, j’ai indiqué dès ma prise de fonctions qu’il était impensable de revivre les tensions du printemps dernier. Le nouveau directeur de l’établissement a adopté des mesures strictes et inédites, qui marquent un tournant dans la gestion des incidents sur le campus concerné. Les quatre étudiants exclus temporairement ont certes été réintégrés, mais après un dialogue très ferme et un avertissement clair sur les mesures qui seraient prises en cas de récidive. Je tiens à le rappeler, la section disciplinaire de Sciences Po Paris reste saisie de ces quatre cas, puisque c’est elle qui est compétente. Enfin, mon engagement politique en faveur de nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche

En deux annonces, Auchan et Michelin ont brutalement acté la disparition de plus de 3 600 emplois. Je veux ici exprimer, au nom de notre groupe, notre totale solidarité avec les salariés et leurs familles. Car oui, une entreprise, une usine, c’est avant tout une grande communauté humaine, qui ne se gère pas avec un tableau Excel. Excel. Pour Michelin, les fermetures des usines de Cholet et de Vannes illustrent la déprise industrielle, en totale contradiction avec les discours tonitruants du Président de la République et de ses gouvernements successifs, rétrofités ou non. J’ai échangé hier, sur le site sexagénaire de Vannes, avec la direction et les représentants des salariés. Je peux témoigner du désarroi, de l’incompréhension et de la colère de ces derniers : ils n’ont eu de cesse de fournir tous les efforts attendus, ils fabriquent des produits qui dégagent des marges, ils permettent à l’entreprise de rémunérer généreusement ses actionnaires,

mais le mal est plus profond. Il prend racine dans le terreau de la naïveté européenne, dans notre décrochage face à une concurrence internationale de plus en plus féroce. Malgré votre politique de l’offre, les défaillances d’entreprises atteignent un niveau record. On dénombre plus de 180 plans de licenciements en France. Tous les territoires et tous les secteurs sont touchés, y compris ceux qui sont liés à la transition énergétique. Nous l’avons entendu, le Gouvernement va enfin demander des comptes au sujet de l’utilisation des aides publiques et proposer un plan de soutien européen à la filière automobile, mais cela ne saurait suffire. Agirez vous enfin pour défendre efficacement les salariés, protéger durablement nos entreprises, nos emplois industriels et notre souveraineté productive, en cohérence avec les objectifs de décarbonation ?

Face à cette situation, notre stratégie et notre politique industrielles doivent reposer sur deux principes. Le premier, c’est de protéger l’existant pour assurer, lorsque les difficultés surviennent,

Les Républicains. Ma question s’adresse à Mme la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Le 30 octobre 2024, en application de la loi de financement

Ce texte sous entend que la majorité des prescriptions de médicaments ne serait pas pertinente, ce qui, vous en conviendrez, madame la ministre, est offensant pour nos confrères et affaiblit leur image.

sont portés sur l’ordonnance ou sur un document dédié […] présenté au pharmacien ou éventuellement à un autre professionnel de santé exécutant la prescription ». Question : si ce document n’existe pas, la prescription sera t elle honorée ? Ce document sera également transmis à la caisse d’assurance maladie. Madame la ministre, du secret médical ? Par ailleurs, alors que l’on parle de déserts médicaux et de la nécessité de redonner du temps médical aux médecins, vous ajoutez une obligation administrative supplémentaire qui ne me semble pas aller dans le sens de la simplification. Madame la ministre, ma question est simple : êtes vous prête à abroger ce décret qui ne fait qu’entraver un temps médical déjà contraint par beaucoup de bureaucratie ?

Ce phénomène se répand, en particulier à cause de la promotion sur les réseaux sociaux de ce type d’usages. Il me semble que l’assurance maladie n’a pas à prendre en charge des produits utilisés en dehors du cadre des indications thérapeutiques.

est probablement beaucoup plus important, hélas ! Le rapport récent du collectif Les Morts de la rue est glaçant. Il met en lumière la mort prématurée de tous ceux qui sont aujourd’hui dans l’ombre. Désormais, ce ne sont plus seulement des publics marginaux qui sont concernés, mais aussi des familles, des femmes, des enfants, comme l’excellent rapport d’information sénatorial sur les femmes sans abri et les travaux de l’Unicef le prouvent. Face à ce constat dramatique, les associations nous alertent : 50 % d’entre elles disparaîtront d’ici à la fin de 2025 si rien ne change. Elles sont le dernier filet de sécurité de notre solidarité nationale, et elles n’ont pas les moyens de faire face. Si elles s’effondrent, c’est le système d’hébergement qui tombe avec elles. Madame la ministre, mieux que personne, vous savez que la crise du logement ne sera pas résolue dans les prochains mois. Pis, la période d’austérité et les crises tant sociales qu’internationales devraient aggraver la précarité dans notre pays. Aussi, madame la ministre, le Gouvernement entend il prendre en compte l’évolution du profil des personnes à la rue réduire le nombre des nuitées hôtelières au profit de places adaptées aux familles et aux enfants ? L’exécutif va t il enfin apporter aux associations un soutien financier fiable, stable et adapté afin d’éviter que nous n’atteignions collectivement un point de non retour ? La parole

Une année s’est écoulée depuis lors et qu’est ce qui a changé ? Rien… La réalité est là : les élus sont toujours autant confrontés aux installations illicites, aux dégradations et, parfois, plus inacceptable encore, aux agressions. Monsieur le ministre de l’intérieur, cela suffit l’Isère, je suis sollicité presque chaque semaine à ce sujet et je n’ai toujours pas de réponses à apporter ; et je crois pouvoir dire que nous sommes nombreux sur ces travées à être dans ce cas. À ces élus, que vais je dire demain ? Que nous déplorons la situation, que nous constatons un problème, mais que nous avons peur et que nous fermons donc les yeux, nous élus, comme les préfets. c’est ce que nous faisons, aujourd’hui, en France, et ce n’est pas acceptable. En réalité, ce qu’il faudrait dire, ce que nous devons dire, à tous nos élus locaux, c’est que nous déplorons cette situation, que nous constatons le problème, mais que nous nous remontons les manches et que nous agissons

Une année s’est écoulée depuis mon élection au Sénat et qu’est ce qui a changé ? Rien, disais je, à une exception près : le ministre auquel je m’adresse Monsieur le ministre, la loi doit être modifiée, c’est une évidence. Il faut donner du pouvoir et des obligations aux préfets, mais aussi des garanties aux maires. Le Sénat est prêt à travailler pour légiférer sur l’accueil des gens du voyage et montrer à nos élus locaux que nous n’accepterons jamais en France que certains soient au dessus des lois de la République Monsieur le ministre, les élus locaux nous donnent un rendez vous et nous ne devons pas le manquer une nouvelle fois. Ici, au Sénat, nous répondrons à leur appel. Nous avons besoin de votre engagement, de votre implication et de votre soutien pour ce travail législatif, qui devra être conclusif. Je compte sur vous ; le Sénat compte sur vous

se passe pas une semaine sans que je sois saisi par un sénateur, une sénatrice, une députée, un député, mais surtout des maires ou des élus locaux, de cette question : l’occupation illicite de terrains publics ou privés par des gens du voyage. Chaque fois, c’est le même scénario, du fait accompli et, bien souvent, celui d’un rapport de force qui s’installe et de l’impuissance des élus ainsi que des forces de l’ordre, lorsque celles ci ne sont pas en nombre suffisant. Bien sûr, cette situation n’a que trop duré. Comprenez moi bien. La République garantit des modes de vie qui peuvent être divers, et je suis respectueux de la liberté et des traditions, mais à condition que l’on respecte les lois de la République ainsi que l’autorité de ceux qui font respecter les lois de la République.

que personne paie la consommation, les dégradations de terrain, y compris d’ailleurs quand les collectivités territoriales mettent à disposition des gens du voyage des aires d’accueil, qui ont coûté très cher. Alors oui, je vous le dis et j’assume,

Ce plan d’action devra désigner une nouvelle doctrine d’intervention des forces de l’ordre – les gendarmes en zone de gendarmerie et les policiers en zone de police – et, surtout, déterminer les dispositions législatives nécessaires,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s’adresse à Mme la ministre du travail et de l’emploi. Madame la ministre, lutter contre la crise de confiance qui affecte le fonctionnement de nos institutions et détourne une partie de nos concitoyens de l’action publique passera, entre autres choses, par le respect des engagements pris et par l’attention portée aux difficultés du quotidien.

Cette volonté du Gouvernement m’avait été réaffirmée en octobre 2023 par la Première ministre, lors d’un déjeuner de travail rassemblant les élus d’outre mer au palais de l’Élysée. Plus d’un an et demi plus tard, la situation n’a pas évolué, elle demeure inchangée. Dans un contexte social toujours extrêmement tendu, marqué par des revendications relatives aux conditions de vie dans ladite outre mer, ce dossier appelle une action sans délai de la part Aussi, madame la ministre, je vous demande de tenir l’engagement pris par votre prédécesseur et je vous invite à saisir le COR dans les meilleurs délais, afin que cette mission soit mise en place dans l’intérêt de nos retraités. Il y va de la plus élémentaire équité, que nous appelons de nos vœux depuis toujours. La parole est

comme vous l’indiquez très justement, les pensions de retraite dans les outre mer sont plus faibles que dans l’Hexagone. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment l’instauration plus tardive des régimes de retraite complémentaires,

dans l’ensemble du pays et, le système étant contributif, le niveau des pensions découle principalement des cotisations versées. Nous appliquons toutefois des mécanismes correctifs,

Pourtant, rien ne se passe aussi simplement que nous l’avions prévu et, dans beaucoup d’endroits, la loi n’est tout simplement pas appliquée. L’État n’applique pas la loi Monsieur le ministre, il s’agit d’un texte simple : deux articles de deux lignes ! Pourtant, une administration, dans une période pendant laquelle le Gouvernement était censé n’expédier que les affaires courantes, a jugé utile de publier une circulaire d’application de huit pages.

Monsieur le ministre, êtes vous prêt à revenir, comme le préconise le Premier ministre Michel Barnier, à plus de simplicité et de bon sens, et à abroger cette circulaire inutile, dans l’intérêt de tous, particulièrement celui des enfants en situation de handicap et de leur famille ?

Je ne vais donc pas faire de langue de bois, je vais vous parler en vérité. Est ce que tout a été bien dimensionné à l’époque pour permettre la mise en place de cette adaptation ? La réponse est non ; j’ai découvert que tout n’avait pas été organisé en conséquence.

M. le ministre délégué chargé de l’industrie. Monsieur le sénateur Jean Michel Arnaud, j’entends évidemment votre préoccupation et je souhaite vous assurer de la pleine mobilisation du Gouvernement pour que les prises en charge des sinistres par les assureurs interviennent rapidement. Le ministre Antoine Armand a encore récemment rappelé à France Assureurs la priorité qui doit être donnée à l’indemnisation des sinistrés, car il est en effet insupportable que des citoyens se trouvent privés de tout et attendent pendant des semaines une indemnisation qui ne vient pas.

remis en application de l’article 52 de la loi organique relative aux lois de finances. La parole est à M.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite ouvrir ce débat sur les finances locales en affirmant avec force, à rebours d’une allégation omniprésente dans le débat public et répandue par plusieurs ministres démissionnaires, que les collectivités territoriales ne sont pas responsables de la situation très dégradée, et même calamiteuse, des comptes publics de notre pays.

peu ou prou à elle seule la dégradation du solde public dans son ensemble. Par contraste, la part des collectivités territoriales dans la dégradation des comptes publics, qui existe, est à relativiser. Certes,

les dépenses des collectivités locales doivent bien augmenter de manière dynamique en 2024, de 4,5 % en fonctionnement et de 13 % en investissement, d’après les dernières informations que nous avons obtenues de la direction générale du Trésor, cette augmentation est essentiellement tirée par le contexte économique et social

Au regard de cet état des lieux, je me réjouis, madame la ministre, du changement de ton de l’exécutif à l’endroit des collectivités territoriales, changement que je retrouve dans vos propos, mais également dans ceux

rappelons que le total des concours financiers de l’État aux collectivités locales est de plus de 50 milliards d’euros. À cet égard, il serait un peu étrange

dont dépend,, ladite santé. Vous l’aurez compris, madame la ministre, je ne conteste pas le principe d’une participation des collectivités au redressement des comptes publics – je le dis avec insistance. Je pense néanmoins que cette participation doit être proportionnée à la contribution des collectivités au déficit et, plus encore, qu’elle doit être équitablement répartie entre elles.

Par la mesure d’assiette, le Gouvernement veut revenir à l’esprit initial du FCTVA, centré sur les dépenses d’investissement. Par la mesure de taux, il veut associer les collectivités à l’effort de redressement des comptes publics. Est ce la bonne façon de faire ? Les collectivités locales sont, je le rappelle, le premier investisseur public, et il ne faudrait pas que la contrainte financière d’aujourd’hui nous pousse à renoncer à des dépenses qui nous permettront de répondre à la contrainte financière de demain.

troisièmement, à la création d’un fonds de réserve des collectivités territoriales, prévue à l’article 64. Sur le papier, un dispositif de ce type ne me paraît pas dénué d’intérêt. Le développement de la péréquation et celui de l’auto assurance collective des administrations locales sont,

que l’architecture globale de ce dispositif me semblent poser de très – trop – nombreuses questions. L’Assemblée nationale, dont je ne commenterai évidemment pas les votes, a purement et simplement rejeté ce dispositif.

Madame la ministre, je conclurai ce propos liminaire par une interrogation. Sous l’égide du président Larcher, un groupe de travail sénatorial a remis l’année dernière un rapport recommandant de réformer dans sa globalité le système de financement des collectivités.

débattre de la situation des finances locales, c’est inévitablement parler de la situation des finances de notre pays. Nous le savons tous, cette situation n’est pas bonne : c’est un fait. En la matière, nous n’avons plus le

dans leur globalité, pour bâtir le juste équilibre que les Français comprendront, car il y va de l’avenir de notre pays. Monsieur le rapporteur général,

à tous les acteurs, citoyens, entreprises, État et collectivités, de participer au rétablissement des finances publiques. Le groupe Les Indépendants veille attentivement au respect, dans ce budget d’urgence,

du taux du fonds de compensation pour la TVA, celui ci passant de 16,4 % à 14,85 %, font craindre le pire pour nos territoires. En effet, le FCTVA permet à nos collectivités d’être partiellement remboursées de la TVA

ci doit en premier lieu moduler ses dépenses de fonctionnement et ne rogner ses dépenses d’investissement qu’en dernier lieu. Les dépenses d’investissement de nos collectivités sont précisément celles qui permettent de financer la transition écologique de nos territoires,

À l’occasion de ce débat, j’appelle votre attention sur une question cruciale pour l’avenir financier de nos départements, à savoir la nécessité d’une augmentation temporaire des droits de mutation à titre onéreux, ces fameux DMTO dont on parle tant. Les DMTO, qui sont des taxes perçues lors de la vente de biens immobiliers,

déjà considérés comme étant « en grande difficulté » en 2024, agissons dès à présent pour les aider à redresser leurs finances. En relevant le taux des DMTO pour une période limitée,

Madame la ministre, nous partageons, vous et moi, deux idées communes : réduire les déficits – il est urgent d’agir – et rendre plus efficiente la dépense publique. le projet de loi de finances pour 2025 me laisse sur ma faim en la matière. Comment se satisfaire d’une simple fusion de Business France et d’Atout France quand il existe encore 400 opérateurs eux tous un budget de 91 milliards d’euros, mais surtout 30 milliards d’euros en frais de fonctionnement ? Pourquoi aborder ce sujet à l’occasion d’un débat sur la situation des finances publiques locales ? La réponse est simple : il faut trouver de nouveaux moyens pour soutenir nos élus locaux dans le financement de leurs investissements indispensables et de leurs services publics. À mon sens, la suppression d’opérateurs pourrait être l’une des solutions. Loin de moi l’idée de faire table rase des opérateurs d’entre eux ont prouvé leur efficacité. En revanche, l’existence d’autres opérateurs est questionnable, pour ne pas dire ubuesque. Comment peut on porter un discours crédible sur l’efficience des dépenses publiques alors que l’État

Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et trois c’est déjà trop. » Imaginez donc à cinq le bazar que ça crée, surtout pour nos élus locaux Madame la ministre, cela m’amène à vous poser cette question : au nom du bon sens, ne faudrait il pas envisager la suppression d’opérateurs dont l’utilité n’est pas démontrée et rediriger les budgets ainsi dégagés vers les collectivités territoriales, en économisant les frais de fonctionnement ?

notamment du fait « d’une épargne brute qui augmente de 9,2 % entre 2022 et 2023 ». Mais, attention, nous savons bien que derrière cette moyenne se cachent de grandes disparités. Comment pourrait on juger de la situation financière du bloc communal en englobant indistinctement le taux d’épargne des grandes métropoles et celui des petites communes ? Si je prends deux indicateurs objectifs de richesse des territoires, le potentiel fiscal et le revenu imposable moyen par habitant, les écarts sont considérables : ils varient du simple au double, voire davantage. Ces écarts nous obligent, me semble t il, à un traitement différencié devant respecter un principe intangible de justice territoriale Or, madame la ministre, parmi les mesures que propose le Gouvernement pour la contribution des collectivités au redressement des comptes publics de la Nation, il y en a une qui me semble particulièrement injuste : la réduction de 2 points du FCTVA, soit une baisse de 10 diminution de recettes toucherait indistinctement toutes les collectivités sans exception et sans distinction de catégorie, de strate démographique ou de richesse. De plus, cette mesure générale réduirait directement la capacité d’investissement des collectivités dans les territoires alors que ces investissements jouent un rôle essentiel dans le soutien aux entreprises locales et à l’emploi. Madame la ministre, pourriez vous reconsidérer cette réduction de 2 points du FCTVA et concentrer les efforts sur des mesures plus justes ?

dans la dette publique est resté stable aux alentours de 9 %, alors que le poids de la dette de l’État sur cette même période a plus que doublé. Dans le même temps, et non sans paradoxe, le Gouvernement s’évertue à imposer des coûts supplémentaires aux collectivités pour réduire le déficit qu’elles auraient creusé.

des cotisations des employeurs publics sans en préciser les contours, sauf pour 2025 où l’augmentation de 4 points est clairement annoncée. Qu’en sera t il pour 2026 et 2027 ?

quant à elle, à +13,48 sur cette même période. Pourriez vous, madame la ministre, apporter une réponse éclairée à tous les employeurs publics ? Doit on s’attendre à une augmentation globale de 13,48 points sur trois ans, ce qui serait une projection insurmontable pour nos services publics

sociale assure les risques vieillesse et invalidité de 2,2 millions d’agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

ce régime pour apporter une réponse concrète. La CNRACL est une caisse qui a fortement contribué, et contribue encore, à l’équilibre d’autres régimes au travers du mécanisme de la compensation démographique. C’est pourquoi j’ai demandé que les mesures visant à élargir la base cotisante pour financer des avantages non contributifs de la branche solidarité vieillesse et de la branche famille

sur notre dette. Avec le changement de gouvernement et la nomination de plusieurs membres de la majorité sénatoriale, on aurait pu espérer sinon des moyens nouveaux dynamiques pour les collectivités, du moins la préservation de leurs ressources. C’est tout le contraire qui s’est produit. Le Gouvernement demande 5 milliards

Après des mois de mise en cause infondée des collectivités locales dans la dérive des finances publiques, communes, intercommunalités, régions et départements sont sommés de contribuer à la réduction d’un déficit qu’ils n’ont pas creusé. L’équilibre budgétaire des départements est préoccupant. Ils subissent déjà un effet de ciseau marqué. La perte de leur levier fiscal, la baisse des DMTO et les transferts de charges – très largement sous compensés – les poussent droit dans le mur. départements sont d’ores et déjà éligibles au fonds de sauvegarde pour 2024. Combien le seront ils en 2025 après contribution ? Alors que leurs dépenses sociales sont en hausse et ne sont pas pilotables, le fonds de précaution prévu par le projet de loi de finances pour 2025

conjugué aux mesures austéritaires de ce budget, conduira à une chute de l’investissement public local et à la fin du soutien porté aux projets des territoires dont les entreprises, les associations et les habitants seront les victimes.

Mes chers collègues, madame la ministre,

et accompagner le développement de nos territoires ruraux comme urbains. Ma conviction est qu’il faut donner tout son sens au partenariat « État collectivités » – je sais que vous y êtes sensible. Cela ne passe ni

Les chiffres sont là : entre 2003 et 2023, les dépenses de personnel des administrations publiques locales ont quasiment doublé, passant de 47,4 milliards par an à 92,6 milliards. Au fil du temps, ni la fusion des régions ni la création des métropoles ou EPCI n’ont permis d’endiguer le phénomène de la hausse des dépenses de fonctionnement et de renforcer l’efficacité des politiques publiques. Ces réformes n’ont fait que multiplier l’addiction et surcharger l’addition. Résultat, on observe que les dépenses des administrations publiques locales évoluent plus rapidement que les dépenses publiques des autres administrations et que le PIB lui même. L’objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement fixé par la loi de programmation des finances publiques pour a été dépassé en 2023 : 5,7 % au lieu des 4,8 % prévus, soit 1,4 milliard d’euros supplémentaires. Ce dépassement est supérieur à l’inflation. La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » J’ajouterai que le meilleur engrais est notre capacité à créer surabondamment de la norme La « fonction » publique est nécessaire, mais elle ne doit pas devenir la « ponction » publique. Il nous faut plus de fonctionnaires territoriaux d’action, mais moins de fonctionnaires d’administrations. Il faut plus de fonctionnaires opérationnels, visibles, au contact du public comme nos pompiers ou policiers municipaux, plus de fonctionnaires au service du pays, moins de fonctionnaires au service de l’État. La responsabilité de ce cercle vicieux n’est pas le fait des élus locaux, qui ne font que répercuter les impulsions parisiennes. Madame la ministre, quelles sont vos propositions structurelles pour endiguer l’emballement des dépenses des administrations publiques locales, tout en retrouvant l’efficacité et en réinsufflant ainsi du consentement à l’impôt ? La parole est à Mme la ministre.

ce volumineux rapport, objet de notre débat, illustre, à lui seul, l’état des relations entre l’État et les collectivités. À l’approche du Congrès des maires, une lecture attentive de cet ouvrage permet de mesurer parfaitement le profond décalage existant entre la théorie et la pratique, entre le verbe et la réalité. S’agissant de la théorie, elle est, comme à l’accoutumée, savamment et adroitement présentée. Et encore, je suis diplomate, car les scandaleuses et mensongères allégations des ministres précédents sur la prétendue responsabilité des collectivités dans le déficit public m’amèneraient à être beaucoup plus cru dans mon expression… Quant au verbe, il s’agit du sempiternel sabir technocratique, triste maquillage d’une réalité devenue malheureusement brutale pour nos collectivités. La réalité et la pratique sont tout autres, madame la ministre Le triste constat c’est que d’une liberté constitutionnelle, pensée et conçue pour garantir la libre administration des collectivités, l’autonomie financière est devenue une coquille vide dépourvue de tout effet utile pour nos collectivités. Le triste constat, c’est qu’en vingt ans le modèle de décentralisation à la française a perdu de sa pertinence face à un double mouvement opéré par l’État consistant à recentraliser le fonctionnement des collectivités locales tout en accroissant, en même temps, les charges pesant sur elles. Dans ce contexte, réconcilier le pouvoir central et le pouvoir local serait une œuvre historique pour la France. C’est même devenu – je le crois sincèrement – un véritable enjeu de démocratie. Y êtes vous prête, madame la ministre ? La parole est à Mme la ministre.

Dans le cas des collectivités locales, par exemple, le Gouvernement a annoncé que celles dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d’euros seront directement concernées par des ponctions sur leurs recettes. Certes, mais selon quels critères précisément ?

madame la ministre, que des communes vont être mises à contribution sans tenir compte des dépenses contraintes ? Tout cela n’est pas des plus judicieux et, sans aller jusqu’à parler de sanction inique, lorsque vous demandez aux collectivités locales de contribuer au redressement des comptes publics à hauteur de 5 milliards d’euros,

votre position sur le versement mobilité additionnel déplafonné, sur la taxe de séjour additionnelle et sur la hausse des péages ferroviaires qui pénalise les régions ? Pouvez vous nous confirmer que la signature de l’État sera honorée s’agissant des

Permettez moi de prendre l’exemple du département du Cher, qui compte 300 000 habitants, mais les difficultés que je décris concernent également de nombreux départements ruraux de taille comparable. Après avoir échangé avec Jacques Fleury, président du conseil départemental, il apparaît que, depuis 2021, le Cher doit faire face à 56 millions d’euros de dépenses supplémentaires, une hausse de 17,5 %, alors que les recettes n’ont augmenté que de 17 millions, une progression de 4,5 %.

dont le Cher, seront dans l’incapacité de présenter un budget en équilibre pour l’année 2025. Ce sera la fin de la cohésion territoriale ! Je rappelle que la dette des départements ne représente que moins de 1 % des 3 200 milliards d’euros de la dette publique ci ne sont pas responsables de la gestion budgétaire du « quoi qu’il en coûte » décidé par le Président de la République. Aujourd’hui, c’est le gouvernement de Michel Barnier qui doit redresser les comptes publics. Dans ce contexte, mes questions sont simples. Quelles mesures concrètes et quels moyens envisagez vous de mettre en œuvre pour que les départements puissent exercer pleinement leurs compétences ? Envisagez vous de mettre en place un partenariat avec les collectivités locales afin de rétablir un lien direct entre fiscalité et démocratie locale ?

N’oublions pas non plus qu’en 2015, sous le gouvernement Valls, ce sont près de 18 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur les collectivités. Peu ont l’air de s’en souvenir ! Surtout à la gauche

et qu’elles ont un rôle déterminant pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique, puisqu’il leur revient d’investir massivement dans la transition écologique, les transports en commun, la rénovation énergétique. De manière générale, les villes portent une grande part de l’investissement public comme du service public. Ce serait donc une folie de sacrifier à ce point leurs recettes de fonctionnement, qui servent aussi à l’autofinancement des investissements.

une dotation globale de fonctionnement égale à zéro et une péréquation qui approche les 800 millions d’euros, la facture de 300 millions, telle

le Gouvernement impose aux collectivités locales une contribution de 5 milliards d’euros – en réalité 9 ou 10 milliards – pour maîtriser le déficit public dès 2025. Or les collectivités locales ont déjà fait beaucoup d’efforts ces dernières années. En 2014, la DGF a fondu de 11 milliards d’euros. En 2018, l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement a été plafonnée à 1,2 % par an. La taxe d’habitation a été supprimée. Pourtant, les collectivités locales font face en première ligne, aux côtés de l’État, à toutes les crises sanitaires, écologiques, énergétiques et économiques, en soutenant le pouvoir d’achat. Dans le même temps, l’État continue de se désengager et les collectivités prennent en charge de plus en plus de missions : la petite enfance, la sécurité, la santé, la transition écologique et le soutien à l’économie à travers leur importante contribution à l’investissement public. Aujourd’hui, elles n’ont plus de marge de manœuvre. Les finances des départements sont exsangues, celles des communes sont fragilisées et les régions sont en difficulté. Or un énième effort est demandé aux collectivités dont le budget de fonctionnement est supérieur à 40 millions d’euros. Elles sont mises à contribution pour alimenter un fonds de précaution de 3 milliards d’euros sans aucune considération de la qualité de leur gestion financière. Dans les Hauts de Seine, cette ponction aveugle atteindrait 102 millions d’euros pour le bloc communal et le département. Madame la ministre, les collectivités locales sont prêtes à participer à l’effort budgétaire national, mais elles souhaitent que leur contribution soit calculée de Dans cette optique et pour tenir compte de la bonne gestion, pourriez vous envisager de remplacer le critère du volume de dépenses de fonctionnement par un critère plus dynamique, celui de l’évolution des dépenses de fonctionnement ? La parole est à Mme la ministre.

la ponction des 6,5 milliards d’euros sur les collectivités locales, déjà fragilisées par la baisse des dotations de l’État depuis de nombreuses années – n’oublions pas l’effet cumulatif de toutes ces mesures –, n’est pas acceptable. Face à leur situation budgétaire détériorée, il nous faut trouver de nouveaux leviers pour financer les investissements des collectivités. Celles ci ont conforté, ces dernières années, leur place de premier investisseur public, à hauteur de 58 % du total. Leurs dépenses d’équipement représentaient 54 milliards en 2022, le bloc communal en portant les deux tiers. Or la suppression totale de la taxe d’habitation en 2023 représente plus de 20 milliards de recettes perdues. Si le débat – relancé… – sur un retour de la taxe d’habitation, quelle qu’en soit l’appellation, a peu de chances d’aboutir, nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il est urgent de redonner aux communes un pouvoir d’agir et une meilleure maîtrise de leurs recettes. Il n’y a pas d’autonomie de gestion sans autonomie fiscale ! Il nous faut redonner des marges de manœuvre fiscale aux communes et retrouver un lien fiscal sur le territoire avec tous nos concitoyens.

Mes chers collègues, madame la ministre,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il me revient de clore ce débat sur la situation des finances locales. Tous les groupes de notre assemblée ont pu s’exprimer, ainsi que les représentants de la commission des finances et le Gouvernement. Je crois pouvoir dire, une fois de plus, que l’exercice a été utile,

21,9 % en 2023 et 13 % annoncés en 2024 – y est pour beaucoup, comme l’augmentation importante de leurs dépenses contraintes, notamment les dépenses afférentes aux allocations individuelles de solidarité, ou encore les dépenses de l’aide

Outre que cette mesure risquerait d’avoir pour effet une diminution de l’investissement local, qui est indispensable autant pour soutenir le tissu économique des territoires que pour relever le défi de la transition écologique, il me semble qu’elle a le défaut majeur de faire dépendre de plus en plus de décisions d’investissement des collectivités de l’accord préalable de l’État. Or l’État peut soutenir tel projet, mais pas tel autre, au moyen de diverses dotations d’investissement. Un maire doit pouvoir mettre ses projets en œuvre sans attendre systématiquement que l’État lui accorde un financement. Enfin, un consensus semble se dégager sur les multiples problèmes que pose le fonds de réserve prévu à l’article 64 du projet de loi de finances, sans qu’une réponse satisfaisante nous soit, à ce stade, apportée pour en modifier la portée. Dans cette conclusion, qu’il me soit aussi permis de verser ma propre contribution à ce dossier complexe et passionnant de la relation entre l’État Pourquoi, finalement, sommes nous ici aujourd’hui à débattre de la juste contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics ? D’où vient le déficit public auquel nous sommes confrontés ? Pas des collectivités locales, nous en sommes tous d’accord. À titre personnel, je pense que la situation actuelle traduit d’abord l’échec d’une politique, qui a été celle des dernières mandatures et qui a notamment consisté à réduire les impôts sans prendre l’élémentaire précaution de réduire en parallèle les dépenses ou de s’assurer d’avoir une croissance suffisante. Ainsi, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, et surtout le maintien de cette mesure en période de crise, constitue à mon sens le péché originel par excellence.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à poursuivre l’expérimentation relative au

Alors que le Sénat examine la présente proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale sur l’initiative du député Nicolas Turquois, je tiens tout d’abord à rappeler combien l’ambition ayant présidé à la mise en place du CDI employabilité (CDIE) est louable : ramener vers l’emploi les publics qui en sont les plus éloignés. Même si le taux de chômage a considérablement baissé depuis 2017, le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour permettre à chacun d’avoir accès à un emploi et à une formation dans un impératif de justice sociale. C’est un enjeu particulièrement brûlant pour les jeunes, les seniors, les moins diplômés de nos concitoyens, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi de longue durée. Le Gouvernement est particulièrement ouvert et attentif – et il restera – à toutes les propositions formulées par le Parlement et qui permettront d’avancer vers l’objectif du plein emploi, sans sacrifier l’impératif de fournir un « bon emploi Le CDIE est porté par des acteurs de l’insertion par l’emploi, dont je sais l’engagement. Il se veut une réponse à ce défi, en sécurisant le parcours professionnel grâce à une embauche en CDI d’un genre particulier. Si les conditions de recours à ce type de contrat sont assouplies par rapport à l’intérim, c’est que l’entreprise de travail à temps partagé (ETTP) est tenue de mettre en place les conditions d’une montée en qualification du salarié recruté en CDIE afin de lui assurer une insertion pérenne dans l’emploi. La promesse de faciliter l’accès à l’emploi stable et durable, que le contrat à durée indéterminée continue d’incarner dans notre modèle social, doit être tenue. Toutefois, nous devons rester prudents pour garantir que le CDIE réponde bien aux objectifs pour lesquels il a été mis en place. À ce jour, avec 5 000 contrats signés depuis 2018 et le début de l’expérimentation, d’après l’inspection générale des affaires

Il était donc important d’avoir un débat éclairé au Sénat à partir des premiers retours d’expérience que nous possédions. C’est ce souci de transparence qui a justifié la transmission au Sénat du rapport d’étape de l’Igas. La première conclusion de l’inspection est précisément la difficulté à réaliser un exercice d’évaluation robuste, alors que les données manquent. Comme le souligne fort à propos Mme le rapporteur, Frédérique Puissat, « l’absence de déclaration des CDIE dans la déclaration sociale nominative (DSN) fait obstacle à une Nous nous engageons auprès de vous, mesdames, messieurs les sénateurs, à créer ensemble les conditions d’un suivi efficace de cette expérimentation. Dans ce cadre, le Gouvernement souhaite qu’une attention toute particulière soit portée aux conditions de travail des des travailleurs en CDIE et à la réalité des contreparties sociales que la loi met à la charge des ETTP qui les emploient. En ce qui concerne les craintes liées à un ciblage trop large des publics éligibles, dont se sont fait écho les auteurs

le dispositif a été recalibré pour répondre à son ambition de ciblage des publics les plus vulnérables. En restreignant l’accès au dispositif et en ciblant davantage les publics, vous répondez aux craintes exprimées de voir ce contrat concurrencer d’autres types de contrats, tels que le CDI intérimaire, dont les titulaires pouvaient répondre aux mêmes critères d’éligibilité. Je crois moi même aux solutions concrètes éprouvées aux réalités du terrain et répondant aux besoins de nos concitoyens. Prolonger l’expérimentation, dont la démarche vise à prouver l’efficacité d’un dispositif avant de le généraliser, si ses résultats sont probants, est le bon choix. La durée de quatre ans apparaît opportune pour garantir le recueil d’un nombre de données suffisant. C’est un préalable indispensable, afin d’avoir le retour d’expérience objectif pour décider ou non d’une généralisation.

Le Gouvernement ne souhaite en effet aucune concurrence déloyale. Il veut seulement engager une action résolue et collective en faveur de l’emploi. C’est pourquoi je me félicite, j’y insiste, que nous puissions nous donner les moyens de prolonger et d’évaluer, avec toute la rigueur qui s’impose, l’expérimentation du CDIE dans les meilleures conditions. Je souhaite toutefois que nous soyons collectivement vigilants et que nous suivions de près durant cette période l’évolution du dispositif et le développement d’éventuels effets de concurrence entre les différents types de contrats. Madame le rapporteur, je vous remercie de votre travail. Vous avez pris en considération les positions et arguments des uns et des autres, sans trahir l’esprit initial du texte ni renoncer à l’attention toute particulière que vous souhaitez porter aux jeunes les moins qualifiés et aux seniors. Mesdames, messieurs les sénateurs, soyez assurés de l’engagement du Gouvernement pour le plein emploi, pour l’accès de chacun à un « bon emploi », qui soit à la fois stable, rémunérateur et de qualité. Je sais pouvoir compter sur votre engagement en la matière. La

Madame la présidente, madame la ministre, madame la vice présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues,

Permettez moi tout d’abord de présenter brièvement la chronologie et le cadre du dispositif. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé, à titre expérimental, le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, le CDIE. Ce dispositif s’adresse à un public spécifique rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle. Ces difficultés sont appréciées selon des critères de substitution définis dans la loi bénéfice d’un minimum social, inscription à Pôle emploi depuis au moins six mois, situation de handicap, âge de plus de 50 ans ou niveau de formation infrabac. Ce dispositif est adossé au régime du travail à temps partagé existant depuis 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

L’expérimentation assouplit en revanche les conditions de mise à disposition en contrepartie des critères restreignant l’éligibilité au dispositif. En effet, la finalité de ce contrat est de s’adresser à un public plus éloigné de l’emploi que la moyenne. Dès lors, l’ETTP est tenue d’encourager la montée en qualification de ses salariés en vue de leur insertion pérenne dans l’emploi. L’entreprise doit, d’une part, leur proposer des actions de formation conduisant à une certification professionnelle, et, d’autre part, abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. Initialement caduque au 1 janvier 2022, cette expérimentation a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi du 14 décembre 2020, pour tenir compte de la crise sanitaire. Voilà donc maintenant dix mois

L’entreprise utilisatrice peut y avoir recours sans avoir à démontrer le caractère temporaire du besoin de main d’œuvre et sans que la durée de la mission accomplie ni les renouvellements soient limités dans le temps. Le secteur de l’intérim dénonce donc une situation inéquitable, une assertion sur laquelle je reviendrai. De même, l’évaluation de l’expérimentation a connu des rebondissements jusqu’à la veille de l’examen en commission. Un premier rapport intermédiaire a bien été remis au Parlement dès 2022. En revanche, l’évaluation finale par l’Igas, produite en juillet 2023, n’a été rendue publique que le 25 octobre 2024. Il faut le reconnaître, rares sont les rapports administratifs ayant suscité autant d’attente. Mais reprenons le fil du texte. L’article 1, adopté par la commission, prévoit une relance de l’expérimentation pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de ce texte. il prévoit de mieux cibler les publics éloignés de l’emploi en resserrant les conditions d’éligibilité. L’accès au CDIE pour les bénéficiaires des minima sociaux ou les personnes en situation de handicap reste inchangé. En revanche, les demandeurs d’emploi devront être inscrits sur les listes de France Travail depuis au moins douze mois, contre six mois auparavant. Cette durée de six mois demeure cependant pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de 55 ans, ainsi que pour les jeunes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur au bac. La commission a également jugé bienvenu l’article 1, qui qui propose de renforcer les droits des salariés embauchés par une entreprise utilisatrice à l’issue d’une mise à disposition dans le cadre d’un contrat de travail à temps partagé, tel que le CDIE. Dans cette situation, ces salariés pourraient rompre leur CDI sans préavis. Par ailleurs, la durée des missions préalablement accomplies dans l’entreprise serait prise en compte, dans une limite de trois mois, pour le calcul de l’ancienneté et pour la période d’essai. Ces droits permettent d’aligner le régime de mise à disposition du travail à temps partagé sur celui applicable au CDI intérimaire. Selon les entreprises du secteur du CDIE, environ la moitié des salariés sont embauchés par l’entreprise utilisatrice à la suite de leur contrat de mission. Cet article de sécurisation va donc dans le bon sens. Au terme de ses travaux, la commission a soutenu le dispositif et adopté sans modification la proposition de loi. Le profil des salariés bénéficiaires a fait l’objet d’attentions particulières de notre part. Est il ciblé sur les salariés les plus éloignés de l’emploi ? D’après les chiffres communiqués par la direction générale du travail, la réponse est oui : 80 % des salariés en CDIE y étaient éligibles au titre de leur inscription sur les listes de Pôle emploi ou de leur niveau de diplôme inférieur au baccalauréat. Les difficultés d’insertion de ce public ne sont pas à démontrer, et le texte resserre encore les critères d’éligibilité en portant à douze mois la condition d’inscription sur les listes de France Travail. Ce meilleur ciblage répond d’ailleurs aux écueils soulevés par le rapport de l’Igas, dont j’ai déjà parlé. Par ailleurs, les ETTP sont soupçonnées de faire une concurrence déloyale au secteur intérimaire, puisqu’elles ne se verraient pas imposer les mêmes obligations légales. Le chiffre de 12 % de différence de coût sur la masse salariale circule, sans qu’il soit sourcé. Après expertise, il correspond en réalité à une différence de modèle d’entreprise, dans la mesure où les entreprises intérimaires mutualisent le financement des périodes d’intermission, là où les ETTP sont tenues légalement d’assurer elles mêmes le salaire horaire de la dernière mission du salarié, ce qui représente, dans la majorité des cas, plus que le salaire minimum prévu dans le cas de l’intérim. En somme, nous avons entendu les inquiétudes, parfois légitimes, que suscitait le CDIE, mais nous pensons qu’un travail de bonne foi des parties prenantes peut dissiper les réserves qui demeurent. Il convient, dans le nouveau régime expérimental créé, de rester vigilant, tant sur son déploiement par les ETTP que sur l’accompagnement des services de l’État. Une première perspective consisterait à établir une convention collective de branche pour le secteur du travail à temps partagé ou, à défaut, à le raccrocher à une branche existante. Dans l’attente, cela ne signifie pas que les salariés en CDIE ne bénéficient pas d’actions en matière de prévoyance ou d’abondement supplémentaire en faveur de la formation. Cependant, ces garanties relèvent d’accords d’entreprise et sont donc moins homogènes, ce qui pose des difficultés, madame la ministre ; nous aurons l’occasion d’y revenir au cours des débats.

Afin de parvenir à ces deux évolutions, les partenaires sociaux doivent se mettre à la table des négociations, mais un accompagnement par les services de l’État est également souhaitable. De même, les services déconcentrés de l’État devront assurer un suivi statistique robuste et un contrôle précis des ETTP, afin de permettre une meilleure évaluation au terme de l’expérimentation. Pour conclure, le CDIE me semble une mesure novatrice pour un public fragilisé sur le marché du travail. Il offre des souplesses aux entreprises dans un environnement économique incertain incertain et permet d’éviter le risque de permittence des personnes les plus éloignées de l’emploi. Il conviendra par ailleurs de nous pencher sur le CDI intérimaire – j’y reviendrai lors de la discussion des amendements –, ainsi que sur les difficultés juridiques que le secteur rencontre, mais c’est un autre sujet que nous aborderons également tout à l’heure.

Madame la présidente, madame la ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, s’il y a un objectif que chacun d’entre nous partage sur ces travées, c’est bien celui du plein emploi. Quelle que soit notre sensibilité politique, nous sommes tous convaincus de la nécessité d’agir, pour permettre à ceux qui ont perdu leur place dans la société de la retrouver par le travail. C’est tout particulièrement le cas des personnes en situation de rupture, d’échec ou de découragement, à qui nous devons donner les moyens de se reconstruire et de retrouver une place sur un marché du travail qui continue de receler des potentialités.

pertinent à cet égard. Fruit d’une initiative parlementaire, ce type de contrat a été créé en 2018 pour relever le défi des contrats précaires, qui touchent actuellement plus de 3 millions de nos compatriotes, plongés dans l’insécurité professionnelle et l’incertitude. Ce dispositif s’impose comme une solution tout aussi bénéfique pour les employeurs engagés dans le travail à temps partagé que pour les salariés qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle et ont des carrières fragmentées. Pour les entreprises, il offre une solution de rechange à l’intérim, tout en permettant de disposer de compétences sur une durée plus étendue. En optant pour ce contrat, les entreprises peuvent mutualiser des ressources humaines et optimiser ainsi la gestion de leur main d’œuvre de manière flexible et efficace. Pour les salariés, souvent confrontés à des réalités professionnelles précaires, le CDIE représente la stabilité tant attendue. En leur offrant des droits comparables à ceux des salariés en insertion durable, il met fin à l’insécurité financière et leur permet d’accéder à une mutuelle, aux congés payés, au crédit et au logement. Loin d’être une faveur accordée aux entreprises qui l’utilisent, ce contrat est la preuve que l’on peut concilier flexibilité et sécurité. En 2010, lorsque j’étais député européen, député européen, j’ai publié un rapport sur la flexisécurité en Europe. J’avais été frappée à l’époque par le retard pris par notre pays pour trouver le juste équilibre entre sécurité et flexibilité du marché du travail. En France, nous avons cette fâcheuse tendance à faire beaucoup de sécurité et à oublier l’indispensable flexibilité, dont nos entreprises ont pourtant besoin. Ce sujet était encore récemment au cœur de nos débats lors de l’examen du projet de loi pour le plein emploi, dont j’étais rapporteur. Cette flexibilité n’empêche pas, on le voit ici, l’octroi aux salariés de garanties, qui sont d’ailleurs renforcées dans la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, avec, d’une part, la possibilité pour le salarié de rompre son contrat de travail à temps partagé sans préavis si l’embauche dans l’entreprise se fait à l’issue d’une mission et, d’autre part, la prise en compte de la durée des missions précédentes pour le calcul de l’ancienneté du salarié. L’intérêt principal de cette proposition de loi est qu’elle vise à mieux cibler les publics éloignés de l’emploi en resserrant les conditions d’éligibilité, ce qui vient renforcer la philosophie sociale du dispositif. En effet, le ciblage des publics défini à l’origine par la loi est aujourd’hui trop large pour atteindre les personnes réellement éloignées de l’emploi. Tout comme notre rapporteur Frédérique Puissat, permettez moi de regretter le manque de réactivité du gouvernement précédent sur ce dossier : absence de transmission au Parlement du second rapport d’évaluation, publication du rapport de l’Igas trop tardive. Résultat, depuis onze mois, plus aucun CDIE ne peut être conclu, faute de prolongation de l’expérimentation. Parce qu’il est nécessaire de ne plus perdre de temps, la commission des affaires sociales a voulu faire preuve de sagesse en adoptant un texte sans modification, même si nous considérons que le dispositif reste perfectible. Là encore, je rejoins Mme le rapporteur sur la nécessité d’un meilleur suivi statistique des CDIE, afin de pouvoir évaluer le dispositif de manière indiscutable. Madame la ministre, vous venez d’ailleurs de vous engager sur ce point. Veillons toutefois à ne pas charger la barque des acteurs de l’emploi, comme France Travail, qui sont trop souvent submergés par ces tâches de collecte. Le temps passé à ce travail administratif, c’est autant de temps en moins pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Quant au périmètre du CDIE, il conviendrait d’encourager certains acteurs de l’emploi à s’en emparer, à l’image des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq), qui jouent un rôle essentiel pour révéler le potentiel des personnes connaissant des difficultés d’accès à l’emploi. Je suis également favorable au rattachement des entreprises de travail à temps partagé à une convention collective de branche professionnelle. Il me semble important de confier aux partenaires sociaux la négociation des modalités de mise en œuvre de ce dispositif

CDI apprenant, CDI intermittent, CDD d’insertion, CDI intérimaire, portage salarial, groupements d’employeurs, travail à temps partagé, prêt de main d’œuvre, travailleurs de plateformes, et Comme le faisait remarquer à juste titre l’Igas dans son rapport de 2023, cette dispersion est source de flou et de complexité pour les salariés comme pour les employeurs, ce qui risque de limiter la portée et l’efficacité Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous sommes favorables à une prolongation de l’expérimentation du CDIE, parce que nous croyons qu’il est nécessaire d’investir dans un avenir où le travail contribue à l’épanouissement personnel et à la justice sociale. Tant de fois j’ai rencontré des personnes au parcours chaotique, pour qui tout semblait perdu, mais qui ont trouvé une vocation, appris un métier et identifié un milieu de travail dans lequel elles s’épanouissent et apportent leur contribution à la société !

telles que celles des lycées professionnels, de l’assurance chômage, ou encore de France Travail, avec pour seul objectif le plein emploi. Les résultats obtenus sont incontestables, avec la baisse de près de deux points du taux de chômage et même une baisse record chez les jeunes. Agir pour le plein emploi, c’est également agir pour ceux qui demeurent les plus éloignés de l’emploi. C’est à cette fin que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 a introduit dans notre droit, à titre expérimental, le contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité. CDIE est destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qu’elles soient en situation de chômage de longue durée, qu’elles bénéficient des minima sociaux, qu’elles soient peu ou pas diplômées, ou en situation de handicap. Le CDIE a un double intérêt : d’une part il offre plus de souplesse à l’entreprise utilisatrice que le CDI intérimaire, celle ci pouvant y avoir recours sans limite de temps et sans avoir à justifier d’un quelconque motif de recours

L’expérimentation du déploiement du CDIE étant arrivée à son terme le 31 décembre dernier sans que nous ait été donnée l’occasion de juger réellement de son efficacité, il nous appartient de considérer la suite. Les données concernant cette expérimentation sont malheureusement très incomplètes, comme cela a été souligné. Environ 5 000 CDIE auraient été signés depuis l’entrée en vigueur du dispositif, dont 1 500 seraient en cours. L’inspection générale des affaires sociales a réalisé une mission d’évaluation de l’expérimentation du dispositif. Ses conclusions, très critiques vis à vis de celui ci, ont été publiées il y a seulement quelques jours, le 25 octobre dernier. L’Igas juge en effet que ce dispositif est resté trop confidentiel et mal connu des différents acteurs. Elle estime qu’il a pu faire l’objet d’un usage détourné par de nombreuses entreprises. Les inspecteurs généraux doutent par ailleurs que le CDIE, dans sa forme initiale, parvienne réellement à assurer « l’employabilité de personnes ayant des difficultés d’insertion Néanmoins, nous estimons que ces conclusions sont particulièrement sévères, au regard du fait que le déploiement du CDIE a été entravé par la crise sanitaire. Les données parcellaires dont nous disposons plaident selon nous pour une évaluation plus approfondie, c’est à dire, concrètement, pour une réactivation de cette expérimentation. Nous pouvons malgré cela constater que le dispositif a d’ores et déjà rempli une bonne part de ses objectifs. Près de 80 % des titulaires d’un CDIE étaient auparavant inscrits à France Travail depuis au moins six mois présentaient, au moment de leur embauche, un niveau de formation égal ou inférieur au CAP ou au BEP. De plus, près de 46 % de ces salariés ont été embauchés en CDI à l’issue de leur mission dans l’entreprise utilisatrice.

En cas d’embauche en CDI par une entreprise utilisatrice du CDIE, le salarié concerné bénéficierait d’une dispense de préavis, de même que de la prise en compte d’une partie de son ancienneté. Nous nous félicitons de ces apports, qui vont dans le sens d’une plus grande sécurisation de ce type de contrat. Parce que nous sommes animés de la conviction que nul ne doit être laissé au bord du chemin de l’insertion professionnelle, nous appelons à poursuivre l’expérimentation de ce dispositif

nous sommes réunis cet après midi pour examiner la proposition de loi visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité. Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité a été créé, à titre expérimental, en 2018, dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Censée prendre fin le 31 décembre 2021, l’expérimentation a été reconduite jusqu’à la fin de 2023 par la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique. Cette variante du CDI classique s’adresse à un public rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle. Pour bénéficier d’un CDIE, il faut répondre à au moins un des cinq critères préétablis,

Factuellement, le CDIE offre plusieurs garanties aux salariés : l’employeur doit notamment prévoir des actions de formation certifiante régulières pour le salarié et abonder son CPF de 500 euros supplémentaires pour chaque année de présence d’un salarié à temps complet. outre, les salariés bénéficiant d’un CDIE sont obligatoirement rémunérés pendant leurs périodes d’intermission, à hauteur de leur dernier salaire horaire de base. Du côté des entreprises, l’employeur n’a pas besoin d’un motif particulier pour recourir au CDIE ; en outre, ni la durée des missions accomplies pour le compte de l’entreprise utilisatrice ni le nombre de renouvellements ne sont limités par la loi, ce qui met tout de même en évidence l’aspect précaire de ce dispositif pour le salarié. En effet, l’absence de limites posées aux renouvellements contribue automatiquement à un rapport de force nettement déséquilibré en défaveur du salarié dans les moments de négociation.

Toutes ces craintes ont été constatées par l’inspection générale des affaires sociales, dans son rapport d’évaluation de juillet 2023. L’Igas l’écrit noir sur blanc : « Le principal intérêt du CDIE pour les entreprises utilisatrices est la grande flexibilité de la mobilisation de la main d’œuvre. Le CDIE est un moyen privilégié de faire travailler des salariés sans limite de temps, tout en conservant la possibilité de s’en séparer quand elles le souhaitent. » Si le groupe du RDSE salue les intentions des partisans de ce dispositif, nous craignons néanmoins qu’il n’ait l’effet inverse de celui qui est À notre sens, faire évoluer des personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle dans un environnement de travail insécurisant n’est pas judicieux au regard de la multiplicité des entraves qu’elles doivent par ailleurs surmonter. Aussi, de manière générale, les experts de l’Igas soulignent qu’il n’est pas établi que le CDIE permette d’atteindre l’objectif qui lui a été assigné, à savoir améliorer l’employabilité de salariés éloignés de l’emploi.

Aussi, dans la mesure où le dispositif a été recentré en tenant compte des recommandations de la mission flash menée par l’Assemblée nationale et du rapport de l’Igas, le groupe du RDSE est plutôt ouvert à donner une nouvelle chance à cette expérimentation. La parole

Toutefois, le CDIE ne s’adresse pas au même public, puisqu’il vise des personnes plus éloignées de l’emploi. De plus, l’ETTP accompagne son collaborateur pour que celui ci améliore ses qualifications et puisse, à terme, jouir d’une meilleure insertion professionnelle. Notre collègue député Nicolas Turquois avait déposé la présente proposition de loi afin de pérenniser ce dispositif. Toutefois, après les auditions qu’il a menées en qualité de rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, il a considéré qu’il était préférable de simplement prolonger l’expérimentation. En effet, la mise en œuvre de ce dispositif a été contrariée, dès le début, par la crise de la covid 19, puis sa montée en charge a été plutôt lente ; on parle de 5 000 contrats conclus entre 2018 et 2023. Dès lors, nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour conclure à la pérennisation du dispositif.

plus pertinent et robuste. Nous regrettons que notre rapporteur n’ait pas eu communication du rapport de l’Igas avant le début de l’examen de la proposition de loi par notre commission.

Enfin, et surtout, les critères d’éligibilité au dispositif ont été revus pour le recentrer sur les personnes rencontrant effectivement des difficultés particulières d’insertion professionnelle.

d’un niveau inférieur au baccalauréat et être inscrit sur cette liste depuis au moins six mois ; être bénéficiaire de minima sociaux ; enfin, être une personne handicapée. J’ajoute que l’article 1, dans sa rédaction issue des travaux en séance publique de l’Assemblée nationale,

Par ailleurs, le texte garantit la reprise de l’ancienneté d’un salarié au titre des missions effectuées dans l’entreprise utilisatrice. Pour conclure, puisque les contours de cette nouvelle expérimentation sont sécurisés

de l’expérimentation, pour quatre années supplémentaires. En juillet 2023, l’inspection générale des affaires sociales a rédigé un rapport d’évaluation du CDIE. Notons qu’il aura fallu attendre le 25 octobre dernier, soit un an et demi, pour que le Gouvernement autorise la publication de cette étude, pourtant essentielle aux parlementaires pour voter la loi. À la lecture du rapport, on comprend mieux pourquoi le Gouvernement a fait le choix de cette rétention d’information. Citons ce document : « Cinq ans après son inscription dans la loi, le CDIE demeure confidentiel : la mission a pu identifier environ 5 000 contrats signés depuis 2018, 2018, dont environ 1 500 en cours, sans garantie d’exhaustivité. En tout état de cause, le dispositif est peu connu des services déconcentrés de l’État, des acteurs en charge de l’insertion sur le terrain et même des salariés concernés, qui le confondent parfois avec le CDI intérimaire. « D’après les investigations de la mission, le CDIE n’est pas utilisé dans un objectif de mutualisation de l’emploi entre plusieurs entreprises, comme c’était prévu, « mais très majoritairement dans un objectif de mise à disposition de salariés auprès d’une seule entreprise, pour des missions de durée en moyenne plus longue que dans le cas de l’intérim classique, voire du CDI intérimaire l’Igas pour décrire ce que nous dénonçons depuis le début, car ce CDI au rabais exclut les travailleurs des protections inscrites dans les conventions collectives, des outils de participation et des avantages du CSE. En effet, le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité a été détourné de son objectif initial, qui visait des travailleurs qualifiés ; il est désormais un outil d’insertion professionnelle pour les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de minima sociaux, les salariés dits peu peu qualifiés, ou encore les personnes en situation de handicap. En dépit des proclamations, le CDIE concerne surtout des ouvriers qui ont traversé une période de chômage. On ne voit pourtant pas pourquoi il faudrait leur proposer autre chose qu’un CDI

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

tous les partenaires ! – s’y opposent. Le rapport commandé par le ministère du travail à l’Igas préconise de ne pas prolonger l’expérimentation et encore moins de la pérenniser, ce qui était votre objectif initial. Vous avez mis ce rapport de l’Igas car il est sans appel. Il dresse un bilan négatif de ce contrat, qui renforce la sédimentation du paysage des contrats de travail. Citons ce document : « Cette dispersion crée un flou et une complexité pour les salariés comme pour les employeurs.

substitue à lui. Sous prétexte de parvenir au plein emploi, on crante chaque fois un contrat plus flexible, en attendant le suivant qui le sera encore davantage. Le CDIE cannibalise ainsi le CDI

sans motif de recours. D’après l’Igas, le CDIE « n’est pas utilisé dans un objectif de mutualisation de l’emploi entre plusieurs entreprises », entreprises, mais très majoritairement dans un objectif de mise à disposition de salariés auprès d’une seule entreprise, pour des missions de durée en moyenne plus longue que dans le cas de l’intérim classique ». En fait, dans la configuration tripartite, les entreprises utilisatrices se désengagent de leur responsabilité sociale d’employeur puisqu’elles ne sont plus parties au contrat de travail, ce qui augmente les risques sociaux liés à l’externalisation de l’emploi. Selon l’Igas encore, « la seule borne à la substitution à l’emploi direct est d’ordre économique, à travers l’arbitrage réalisé par les entreprises utilisatrices au regard du coût relatif de l’externalisation et de l’embauche directe Plus le surcoût du recours au CDIE par rapport à l’embauche directe est modéré, du fait de la baisse des droits des salariés, plus cela conduit à une large substitution à l’embauche directe.

pourrait paradoxalement les enfermer dans une relation triangulaire de travail potentiellement porteuse de risques, et devrait le cas échéant être assortie de garanties conventionnelles supplémentaires ». Le cadre légal du CDIE est

à renforcer le parcours d’insertion d’une population vulnérable. En conclusion, rappelons que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun doit rester le principe ; les contrats de travail atypiques doivent rester l’exception et non se multiplier.

L’objet de cet amendement était d’« expérimenter pendant trois ans un nouveau dispositif de travail à temps partagé, le travail à temps partagé aux fins d’employabilité », en s’appuyant sur les entreprises de travail à temps partagé, les ETTP. pour défendre cette proposition était qu’en 2018 « les dispositions législatives relatives au travail à temps partagé [étaient] en pratique très peu utilisées depuis leur mise en place qui remonte pourtant à de nombreuses années – C’est avec attention que nous avons pris connaissance des arguments des différentes parties prenantes quant à l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité. Nous avons aussi pu lire le rapport de l’Igas

et peut être mis à disposition d’entreprises utilisatrices sans limite de temps et sans avoir à justifier d’un quelconque motif de recours. « Alors que la loi de 2005 cible cette mise à disposition sur du personnel qualifié auprès d’entreprises qui ne peuvent recruter directement “en raison de leur taille ou de leurs moyens”, le CDIE vise quant à lui “des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle”, sans condition sur l’entreprise de mise à disposition. » Si l’Igas souligne que le cadre légal du CDIE est plus avantageux pour le salarié

que, cinq ans après sa création, le succès du CDIE est tout relatif : seuls 5 000 contrats auraient été signés depuis 2018, dont environ 1 500 seraient en cours. Le grand intérêt du CDIE pour les entreprises qui y ont recours serait la grande flexibilité de la mobilisation de la main d’œuvre. Cela contribue à faire du CDIE un contrat présentant un faible risque de requalification. Si l’on peut y voir un atout pour l’entreprise utilisatrice,

Soumises à de moindres obligations légales et conventionnelles, elles ne connaissent pas non plus la contrainte des conventions collectives. C’est dire que les intérêts des salariés ne sont garantis, pour une large part, que par la bonne volonté des ETTP. Si ces dernières semblent avoir fait preuve d’une l’Igas souligne néanmoins « une grande hétérogénéité des pratiques au sein des ETTP ». Par ailleurs, la bonne volonté de ces entreprises constitue un fondement plus fragile que le droit pour asseoir la situation des travailleurs concernés. Selon l’Igas, il serait fait recours au CDIE non pas « dans un objectif de mutualisation de l’emploi entre plusieurs entreprises, mais très majoritairement dans un objectif de mise à disposition de salariés auprès d’une seule entreprise, pour des missions de durée en moyenne plus longue que dans le cas de l’intérim classique des missions de durée fort longue ! L’objectif annoncé dans l’amendement qui a permis la création du CDIE, à savoir favoriser le travail en temps partagé, n’est donc pas atteint. Il est d’ailleurs frappant que de grandes entreprises comme La Poste soient d’excellentes clientes du CDIE, alors qu’elles auraient sans aucun doute les moyens d’embaucher les bénéficiaires de CDIE par le biais de CDI traditionnels, voire de contrats de travail intermittent. Dans ce contexte, le CDIE apparaît comme un moyen pour des acteurs économiques désireux d’avoir une politique salariale et de ressources humaines beaucoup plus souple que ne l’exige le droit du travail. Ils peuvent ainsi officier sans crainte de voir des contrats de travail de court terme requalifiés par la justice. L’Igas estime enfin que le but avoué du CDIE – assurer l’employabilité des personnes éloignées de l’emploi – n’est pas susceptible d’être atteint au vu du fonctionnement du dispositif. Ses critères de recrutement sont en effet trop larges. Il s’appuie aussi sur un doublement de l’abondement du compte personnel de formation. Le CPF ne serait peut être pas le bon outil pour ce faire, et les ETTP n’ont en tout état de cause pas toujours pu assurer cet abondement. Au regard des éléments que nous avons eu à connaître, il apparaît évident que les ETTP ont rempli leur part du travail en ce qui concerne le CDIE. Pour autant, cela ne suffit pas. Rien ne garantit que des acteurs moins scrupuleux ne se saisiront pas de ce dispositif et que les salariés travaillant en CDIE ne resteront pas indéfiniment coincés dans ce statut précaire. Le CDIE est au contraire susceptible d’apparaître comme un coup de canif porté au droit du travail pour satisfaire des politiques managériales discutables. Le droit du travail est un conquis social, qu’il faut en tout état de cause protéger de stratégies visant à le fragiliser en instrumentalisant les travailleurs. Arguer que mieux vaut un travail avec très peu de protections sociales et conventionnelles que pas de travail du tout n’est pas audible. Nous avons déjà entendu ce type d’arguments concernant les travailleurs ubérisés, et nous les avons refusés. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité. Certes, l’Assemblée nationale a recadré le dispositif par voie d’amendement, mais nous considérons qu’il existe suffisamment de solutions dans le domaine de l’insertion par l’économie sans que soit créé un outil supplémentaire qui pourrait être utilisé à des fins non conformes au droit du travail.

Le CDIE, contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, est né, à titre expérimental, avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il s’appuie lui même sur la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dispositif par lequel une entreprise recrute du personnel qualifié, qu’elle met à disposition d’une entreprise utilisatrice pour une mission particulière.

», c’est à dire des personnes de plus de 50 ans, celles dont le niveau de formation est inférieur au bac, les bénéficiaires de minima sociaux, ou encore les personnes en situation de handicap. Ce type de contrat dispense l’entreprise utilisatrice de certaines obligations par rapport au CDI intérimaire, avec lequel on le compare beaucoup. En l’occurrence, elle n’est obligée de prouver ni que son besoin est strictement temporaire ni que la mission proposée est limitée dans le temps. En contrepartie, toutefois, afin que le « E » employabilité – du CDIE soit pleinement justifié, l’entreprise de travail à temps partagé est tenue de proposer aux salariés des actions de formation certifiantes et d’abonder le compte personnel de formation (CPF) des salariés à hauteur de 500 euros supplémentaires par an. Après avoir été renouvelée une fois, l’expérimentation du CDIE est arrivée à son terme le 31 décembre 2023. La proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale visait initialement à pérenniser le dispositif.

Il pointe notamment la faiblesse des données qui en permettraient une évaluation fiable. Cependant, il semble que ce manque de données provienne moins d’une absence de volonté des entreprises de les faire remonter que du manque d’outils adéquats pour y procéder. C’est pourquoi je me réjouis que la proposition de loi, dans sa nouvelle rédaction, vise à prolonger l’expérimentation. Il faudra que ces quatre années supplémentaires permettent de corriger les lacunes et de renforcer la remontée des données. Par ailleurs, le texte vient aussi resserrer le dispositif, pour mieux s’assurer qu’il concerne le public visé. Les demandeurs d’emploi devront être au chômage depuis un an, contre six mois actuellement, et le contrat s’adressera aussi aux personnes de plus de 55 ans, contre 50 ans actuellement, qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins six mois. Enfin, j’estime que le dispositif du CDIE s’inscrit dans la logique de réformes importantes, que le Sénat a votées en 2023 part, la réforme des retraites, qui impliquait nécessairement de mieux accompagner les seniors vers l’emploi, d’autre part, la loi pour le plein emploi, qui visait notamment les bénéficiaires du RSA. Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité nous semble donc aller dans le sens de l’accompagnement vers l’emploi d’un public qui peut en être éloigné. C’est pourquoi le groupe Les Indépendants votera en faveur de la prolongation de son expérimentation.

non conclusif ». En effet, au mépris des obligations de l’article 115 de la loi du 5 septembre 2018, les ETTP contractant des CDIE n’ont remonté que peu de données, de faible qualité, rendant impossible l’évaluation six mois avant la fin de l’expérimentation.

les critiques et les inquiétudes. Le Gouvernement a pris des engagements sur le suivi. Par ailleurs, il faut que ce texte puisse être adopté conforme pour que nous puissions aller vite et poursuivre l’expérimentation dans de bonnes conditions.

[En effet,] le ciblage des publics défini par la loi est trop large pour atteindre les personnes vraiment éloignées de l’emploi et recoupe largement celui des CDI intérimaires ». Par cet amendement, nous entendons restreindre les conditions d’éligibilité pour l’accès au CDIE,

Selon l’Igas, « pour les entreprises utilisatrices, le CDIE répond à un besoin de fidélisation des salariés mis à disposition, mais aussi de flexibilité, sans pour autant s’appuyer sur un cadre juridique adapté » à l’usage de l’intérim. Dans ce rapport, il est indiqué que 6 % des CDIE ne présenteraient aucun des critères d’éligibilité définis par la loi. Enfin, la proposition de loi initiale prévoyait des sanctions. Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a supprimé

Mme Raymonde Poncet Monge. Les salariés en CDIE sont particulièrement vulnérables. Ils ont d’autant plus besoin des droits ouverts par une convention collective pour conforter leur retour vers l’emploi durable.

de branche. Le ministère du travail encourage tous les employeurs à être couverts par un accord de branche, entre autres pour cette raison. En l’absence de toute régulation de branche, et alors même que les droits à formation sont théoriquement doublés, après quatre ans d’expérimentation, les ETTP contractant des des CDIE présentent un bilan de formation professionnelle pauvre, en qualité et en quantité. Comme le soulignent les partenaires syndicaux et patronaux de la branche du travail temporaire, avec ce piètre bilan en termes d’accès à une formation professionnelle qui conditionne le retour à l’emploi durable, le recours aux CDIE relève principalement de l’effet d’aubaine, puisqu’il offre une flexibilité accrue, assorti d’une moindre sécurité pour les salariés. D’ailleurs, selon l’Igas, « construit en dehors du cadre du travail temporaire, le CDIE échappe un encadrement qui vise, en France comme dans de nombreux pays, à limiter les risques sociaux liés à l’externalisation de l’emploi ». Cet amendement de repli vise donc à rendre obligatoire l’ouverture d’une négociation de branche